Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle l'examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'adhésion de la France à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française,

l'amendement n° 186 rectifié. Cet amendement tend à inscrire dans la loi le principe de la prise en compte de la soutenabilité de l'évolution des redevances pour les finances des autorités organisatrices de transport. Une très forte augmentation de redevances, telle que prévue dans le cadre du contrat de performance, peut par exemple paraître incohérente avec la demande émise par l'État quant à la maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement des grandes collectivités. Aussi, cet amendement a pour objet de prévenir toute présomption de soutenabilité des majorations tarifaires pour les services conventionnés. a considéré à plusieurs reprises que la soutenabilité des péages devait faire l'objet d'une appréciation spécifique pour les services conventionnés, dès lors que la capacité du marché à les supporter est biaisée par l'existence d'une subvention publique versée par les

la définition de segments de marché adaptés aux services conventionnés devrait déjà permettre d'apprécier correctement la soutenabilité des redevances pour ces services. les tarifications proposées par SNCF Réseau au cours des dernières années, ainsi que les évolutions du décret encadrant le système tarifaire ne le garantissent pas. Avec ces amendements s'agit d'énoncer expressément, au niveau législatif, la nécessité de prendre en compte les spécificités des services conventionnés par une appréciation adaptée de la soutenabilité des péages et de la capacité du marché

mettaient en péril le développement du fret ferroviaire ou la desserte de tous les territoires par les TGV.

près de trois fois moins vite que les dépenses d'entretien et de régénération du réseau correspondant. Gardons à l'esprit qu'il faut préserver un équilibre global entre les ressources et les besoins : il ne faudrait pas non plus que des baisses de péages se traduisent par des baisses équivalentes de dépenses d'entretien.

vont permettre d'ouvrir le débat. Mais vous devez nous dire où est la garantie que, demain, l'État ne dira pas aux régions : « Puisque c'est vous qui voulez cette ligne-là, c'est vous qui allez payer.

? Cet amendement vise tout simplement à modifier l'importance donnée aux gains de productivité des entreprises ferroviaires pour le calcul des redevances d'infrastructure. Il ne s'agirait plus de « respecter

productivité dans le mode de calcul des péages ? Certains gains de productivité peuvent être dus à l'action du gestionnaire d'infrastructure ; d'autres peuvent être des initiatives de l'opérateur ou d'une rupture technologique. Imaginons qu'une région modernise une ligne, par exemple grâce à un dispositif de commande et de contrôle,

garantir un juste bénéfice des gains de productivité, tant pour l'opérateur et l'autorité organisatrice que pour le gestionnaire d'infrastructure.

d'un document-schéma, le SRADDET, qui prévoit un schéma des mobilités interne aux régions. Nous proposons que ce document permette de déterminer les lignes et dessertes

du système de transport ferroviaire, instance d'information et de concertation des parties prenantes du système de transport ferroviaire national, accomplisse un travail

d'identifier les dessertes dont l'équilibre économique est fragile sans modulation des péages. Des travaux techniques approfondis seraient des principes objectifs de modulation à partir d'études fines relatives à la situation économique des lignes, entre le gestionnaire d'infrastructure et l'ARAFER. À ce stade, il ne nous paraît donc pas judicieux

Par ailleurs, il ne nous semble pas pertinent de soumettre des schémas régionaux au Parlement. Le système de schémas proposé cet amendement nous semble donc complexe et peu adapté aux conditions concrètes de mise en oeuvre de la tarification du réseau ferroviaire.

qui « fixe les orientations de l'État concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national ». Il est également indiqué que ce schéma « détermine, dans un objectif d'aménagement et d'égalité des territoires, les services

Il accorde une attention particulière à la prise en compte des besoins de capacités en matière de fret ferroviaire. Nous souhaitons plus spécifiquement appeler l'attention sur les autoroutes ferroviaires, particulièrement pertinentes en matière de report modal de la route vers le rail pour les longues distances.

Force est en effet de souligner que ces autoroutes ferroviaires sont confrontées à des contraintes de circulation récurrentes qu'il est nécessaire de prendre en compte si l'on souhaite relancer avec quelque chance de réussir le fret ferroviaire. Quel

industrie lourde, est tellement coûteux que c'est le même réseau qui est utilisé dans les deux cas. Pour les opérateurs, il y a quelquefois une

Merci, monsieur le rapporteur

ter La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article. Actuellement, pour le transport ferroviaire de voyageurs, les seules dessertes que peuvent proposer sur le territoire français les opérateurs distincts de SNCF Mobilités sont les dessertes de « cabotage » dans le cadre d'un trajet international. Le présent article, pour acter l'ouverture totale à la concurrence prévue par le projet de loi, pose le principe selon lequel toutes les entreprises ferroviaires, et non plus seulement SNCF Mobilités et les opérateurs de fret ferroviaire, pourront désormais assurer librement des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Cette ouverture est conditionnée à la possibilité pour l'autorité de régulation de limiter ou d'interdire l'exercice de cette « liberté au nom de la préservation de l'équilibre économique des contrats de service public, c'est-à-dire de l'offre de TER et de TET. Il s'agit d'une bien faible limitation dans les faits, puisque le principe est bien celui de la concurrence. Ainsi, demain, n'importe quelle entreprise ferroviaire de n'importe quel pays pourra intervenir sur le réseau de TGV, venant directement concurrencer la SNCF à sa guise sur les trajets de son choix. Il y a fort à parier que, malgré les systèmes d'encadrement et les variations de péage, des pans entiers du territoire seront laissés à l'abandon faute de rentabilité suffisante et donc de prétendants- nous avons beaucoup échangé sur ce sujet

que s'il y a volonté de l'autorité organisatrice de s'en saisir. Il ne faudra plus compter sur la SNCF pour exercer des missions de service public, puisque les outils de péréquation auront été brisés et la SNCF sommée de se comporter comme un opérateur privé. Une telle réforme condamne en réalité le service public ferroviaire et menace gravement le maillage du territoire. Soyons clairs, ce qui pénalise l'offre « grande vitesse », ce n'est pas l'absence d'opérateurs alternatifs, mais la vétusté du réseau, qui entraîne régulièrement une pagaille monstre et des ralentissements sur des kilomètres et des kilomètres de rail. Cette réforme est donc avant tout

article précise les conditions d'ouverture à la concurrence, à partir du 12 décembre 2020, des lignes pour les services librement organisés de transport ferroviaire. Conformément à notre vision globale du service public ferroviaire, nous nous opposons à cette première étape calendaire de son démantèlement. On nous explique que ce pacte ferroviaire va aussi protéger, puisqu'il est question d'introduire un encadrement de ces nouveaux services librement opérés, mais la seule limite posée posée à la concurrence libre et non faussée entre entreprises ferroviaires est l'atteinte à l'équilibre économique des contrats de service public mis en oeuvre soit par les régions, soit par l'État. Pis, cette atteinte devra être constatée par l'ARAFER, à laquelle on donne le rôle d'arbitre, mais qui, comme toute autorité prétendument indépendante, n'a pour fonction que d'accompagner la libéralisation du rail. Pour notre part, nous pensons que c'est à l'État de prendre ses responsabilités en utilisant toutes les possibilités offertes par le règlement OSP de dérogations à l'ouverture à la concurrence pour l'ensemble de l'offre ferroviaire, qu'il soit conventionné ou dit « libre TGV doit être complémentaire de l'offre de TET et de l'offre de TER, et non pas concurrente. Nous prônons un système ferroviaire qui privilégie les complémentarités et les interconnexions qui sont favorables aux usagers. Aujourd'hui, pourront saisir l'ARAFER, les autorités organisatrices, le gestionnaire d'infrastructure ou l'entreprise chargée de l'exécution du contrat. C'est tout de même limité ! Pourquoi ne pas ouvrir ce droit de saisine aux associations d'usagers, aux comités de lignes ? Nous ne sommes pas Nous ne sommes pas convaincus par les expériences étrangères d'ouverture à la concurrence, pas plus que par l'exemple national d'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire, qui

amendement vise à supprimer les dispositifs qui permettent à l'ARAFER de réguler le développement des services librement organisés. Je suis donc un peu surprise que vous n'adhériez pas à ces dispositifs qui permettent de s'assurer que les services librement organisés ne perturbent pas les contrats de service public. L'objectif est de profiter pleinement des opportunités offertes par l'ouverture à la concurrence, et donc des nouveaux services qui peuvent être proposés aux voyageurs, tout en donnant une priorité aux contrats de service public. Il me semble que vous pourriez

puis du transport international en 2010 et, enfin, du transport national de voyageurs aujourd'hui. Nous avons besoin de revenir à un modèle unifié, intégré, faisant l'objet d'un monopole permettant une péréquation entre les différentes activités et qui soit chargé d'une mission de service public claire, dont l'État ne se défausse ni sur les régions ni sur le privé.

et économiques. L'ouverture à la concurrence, elle, n'est absolument pas dictée par l'intérêt général. Parce que se déplacer est une liberté fondamentale dont le droit au transport est un support essentiel, 95 % des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports provenaient l'année dernière du mode routier, parce que le niveau global d'émission de particules fines a encore augmenté cette année, malgré l'accord de Paris, parce que le rail est un transport économique- la pollution de l'air et les accidents corporels issus du mode routier coûtent bien plus à nos sociétés -, parce que les TET, les TER et le fret de proximité sont des facteurs de cohésion et de désenclavement territoriaux et parce que l'industrie ferroviaire est une filière stratégique représentant 4,2 milliards d'euros seul l'intérêt général, auquel on ne peut opposer l'exigence de rentabilité financière, doit guider les choix d'orientation, d'investissement et de gestion des services publics

Nous proposons donc d'en revenir à la définition inscrite dans la LOTI des missions d'un groupe public unifié chargé d'assurer la cohérence de l'ensemble des services intérieurs sur le réseau ferré national. En effet, nous considérons que l'ouverture à la concurrence est le gage d'une complexité nouvelle et d'un risque accru pour la sécurité, comme le montre notamment l'exemple britannique. Je sais que vous n'aimez pas qu'on le cite, mais les faits sont là : le taux d'accident dans très largement progressé depuis l'ouverture à la concurrence. La nature même du réseau exige une gestion cohérente et coordonnée de l'exploitation au niveau national.

et à l'intérêt général. L'existence d'un monopole confié au groupe public ferroviaire a été justifiée il y a quatre-vingts ans, et la création de la SNCF par la nature même du service, que les créateurs ont voulu extraire des règles de marché

pourquoi laisser à la main invisible du marché le choix du maintien de telle ou telle desserte, sans que la cohérence globale de l'offre soit assurée ? C'est incompréhensible ! La nature spécifique de cette mission d'intérêt général a d'ailleurs justifié pour la SNCF le statut d'EPIC, doté de prérogatives de puissance publique. Aujourd'hui, derrière la remise en cause du statut de l'entreprise, puis de celui des cheminots, derrière la libéralisation du rail, se dessine le véritable objectif de votre réforme supprimer toute idée même de service public, en faisant du transport un service purement marchand. Nous pensons, pour notre part, que la maîtrise publique est le meilleur gage d'un service cohérent et performant. C'est pourquoi nous plaidons pour un système d'exploitation unifié et en situation de monopole, un système en mesure de répondre à sa mission d'intérêt général.

à mi-chemin entre nous, la gauche, et nos collègues du groupe Les Républicains ; mais, idéologiquement, vous avez fait le choix de basculer dans le monde du libéralisme. Nous,

à préciser que les entreprises ferroviaires peuvent effectuer des services commerciaux lorsque les autorités organisatrices n'attribuent pas directement des contrats de service public, en application des dérogations à l'obligation de mise en concurrence des services conventionnés prévue par le droit européen.

S'il s'agit d'affirmer la prééminence des services conventionnés attribués sans mise en concurrence, la commission ne peut évidemment pas accepter l'amendement. D'une part, le conventionnement des services publics a pour objet de combler les défaillances du marché et n'a pas vocation à être effectué pour l'ensemble des services ferroviaires. D'autre

enjeux d'aménagement du territoire au travers des différents dispositifs qui figureront dans la loi. Quant aux services conventionnés, ils permettront aux régions

de vote. Nous avons voté le quatrième paquet ferroviaire, adapté en France avec de très nombreuses dérogations obtenues, notamment, par Alain Vidalies. Nous sommes favorables à une maîtrise

l'ARAFER. Dans le cadre de l'article 1 , lorsque la saisine est justifiée pour définir, sur un service librement opéré, une atteinte à un contrat de service public, la saisine est, hélas, extrêmement limitative, puisque réservée à l'autorité organisatrice, à l'opérateur ou à l'État., à l'État., à l'article 2 , lorsqu'il s'agit de l'application par l'autorité organisatrice des exceptions prévues par le règlement OSP, la formulation est permissive, visant « toute toute personne à qui la décision est susceptible de faire grief ». Nous considérons que ce décalage est révélateur : lorsqu'il s'agit de favoriser la concurrence, la saisine est large ; à l'inverse, lorsqu'il s'agit de préserver le service public ou, du moins, la délégation de service public, elle est très encadrée. Cet amendement est un amendement de repli, puisque, sur le fond, nous contestons la libéralisation des services librement organisés- vous l'avez compris, et nous avons compris que c'est un gros point d'achoppement.

saisine de l'autorité administrative compétente, du gestionnaire d'infrastructure ou de l'autorité organisatrice qui a attribué le contrat, ou encore de l'entreprise ferroviaire qui l'exécute. Si nous considérons que le rôle de l'ARAFER est de veiller en tant qu'autorité de régulation au au bon fonctionnement des marchés de service public de transport de voyageurs, nous estimons aussi que l'on ne peut pas laisser cette autorité se prononcer sur la régulation du droit d'accès au réseau sur le fondement de critères visant exclusivement l'équilibre

amendement, nous souhaitons préciser les critères qui seront utilisés par l'ARAFER, afin de définir si une ligne librement exploitée porte atteinte ou non à l'équilibre d'un contrat de service public.

Nous proposons de retenir comme critères d'un test d'équilibre non seulement des éléments financiers et économiques traditionnels, tels que les dispositions relatives à l'équilibre économique prévues par le contrat de service public, les pertes de recettes et coûts supplémentaires éventuels à court et moyen terme, les bénéfices éventuels à court et moyen terme, l'évolution de la rentabilité des services exploités par le titulaire du contrat de service public, mais également des éléments plus généraux relatifs à l'impact environnemental de ces nouvelles liaisons, l'accessibilité financière pour les usagers, ou la cohérence de la liaison projetée par les politiques locales d'aménagement du territoire. Il s'agit, vous l'aurez compris, d'encadrer les pouvoirs confiés ici à l'ARAFER, afin de prendre en compte l'ensemble des inconvénients qui peuvent naître d'une exploitation nouvelle et de garantir ainsi le maintien du service public dans des conditions pérennes. Quel

empêcher l'ARAFER de se prononcer sur un service librement organisé qui pourrait perturber un contrat de service public, même si ce service fait partie du schéma national. Il me semble vraiment qu'il faut donner la priorité au contrat de service public.

font partie des éléments qui sont forcément pris en compte par l'autorité organisatrice dans la définition du contrat de service public. Là encore,

de multiples acteurs du secteur ferroviaire : des représentants des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des grands ports maritimes, des opérateurs de transport combiné de marchandises, des partenaires sociaux, des chargeurs, des voyageurs, des associations de protection de l'environnement agréées, des personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national, ainsi que deux

la mission d'effectuer un suivi des aspects économiques du système de transport ferroviaire, en particulier son ouverture à la concurrence, et à étendre ses compétences. Ainsi, le Haut Comité pourra rendre des avis ou adresser des recommandations au ministre chargé des transports, sur son initiative ou sur saisine de celui-ci. Il pourra également demander des travaux de recherche et des études socio-économiques relevant de son domaine de compétence auprès des organismes placés sous la tutelle des ministres chargés des transports,

des aspects économiques du système de transport ferroviaire et qu'il ait la possibilité de donner un avis sur les modalités d'ouverture à la concurrence, notamment sur la base du rapport de l'ARAFER.

d'autant plus que nous n'avons obtenu ni étude d'impact ni avis du Conseil d'État, et que nous légiférons « au doigt mouillé » sur de nombreux articles que le Gouvernement a lui-même insérés dans le projet de loi initial, qui n'était composé que d'articles d'habilitation à légiférer par ordonnance.

Rien ne garantit non plus que la transformation des EPIC en sociétés anonymes permettra de maintenir, voire de renforcer la qualité du service public. Pour toutes ces raisons, les auteurs de l'amendement considèrent que cette loi ne peut être envisagée, en quelque sorte, sorte, que comme une grande loi d'expérimentation, nécessitant de fixer un rendez-vous au Parlement pour en évaluer tous les effets dans quelques années. Aussi proposons-nous de fixer une clause de revoyure avant la fin de l'année 2023 sous l'égide du Haut Comité du système de transport ferroviaire.

afin de tirer des conclusions sur les éventuelles adaptations qui s'imposeraient. C'est par exemple ce qu'ont fait vos collègues députés Gilles Savary et Bertrand Pancher à l'Assemblée nationale sur la réforme ferroviaire adoptée en 2014.

Créé par la réforme ferroviaire de 2014, ce haut comité a pour mission d'éclairer le Gouvernement et le Parlement sur la situation du système ferroviaire national, ses évolutions envisagées ou prévisibles. Dans ses avis, celui-ci prend en compte tous les aspects juridiques, financiers, économiques, sociaux, environnementaux, afin de proposer ou d'évaluer les grandes orientations de la stratégie nationale dans le domaine ferroviaire. Avec cet amendement, on ne crée donc pas- je le précise bien -de tâches supplémentaires pour ce haut comité, qui remet simplement son rapport au Gouvernement et au Parlement dans les mêmes délais et les mêmes termes. L'ouverture à la concurrence des systèmes ferroviaires a eu des effets variés selon les pays étudiés, certaines expériences se soldant par des échecs et d'autres par des succès. En parallèle, un certain nombre d'études soulignent que l'organisation du travail et le degré d'ouverture à la concurrence ne constitueraient que des éléments paramétriques, le critère fondamental en matière d'augmentation de la qualité de service restant le montant de l'investissement public. Devant ces situations plurielles et contrastées, il apparaît nécessaire d'informer les Français,

en plus, il suffit d'envoyer le rapport à un certain nombre de parlementaires. Vous n'allez pas me répondre que vous n'allez pas soutenir cet amendement ! Sinon, je serai très vexé

des exploitants d'installations de service reliées au réseau ferré national et des autorités organisatrices de transport ferroviaire. C'est au sein de cette instance que SNCF Réseau dialogue avec ses clients, également membres. La vocation de ce lieu d'échanges est d'améliorer les relations, notamment

fournie aux utilisateurs du système de transport ferroviaire national ; préserver la sûreté des personnes et des biens, la sécurité du réseau et des installations relevant du système de transport ferroviaire national ; organiser et piloter la filière industrielle ferroviaire, en vue d'en accroître la capacité à l'exportation, la sécurité, l'efficience économique et environnementale, la fiabilité, le développement technologique, la multimodalité et l'interopérabilité ; programmer les investissements de développement et de renouvellement du réseau ferroviaire ; assurer la complémentarité entre les services de transport ferroviaire à grande vitesse, d'équilibre du territoire et d'intérêt régional, pour satisfaire aux objectifs d'aménagement du territoire. Il nous paraît important, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, d'élargir les missions du comité des opérateurs du réseau et de mettre un peu d'huile dans ses rouages complexes. Quel

peut effectivement jouer un rôle important dans les différents domaines évoqués par l'amendement : cohérence de l'offre proposée aux voyageurs, permanence opérationnelle du système

des transports, tel qu'il résulte de la loi du 4 août 2014, confie à l'État le soin de veiller à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national,

Nous avons au contraire besoin de consolider la valorisation, dans la durée, des salariés au sein de l'entreprise, leurs conditions de travail et leur technicité. La fidélisation du personnel étant un élément déterminant de la qualité du service rendu, la remise en cause du statut

J'espère aussi que nous aurons une convention collective de branche de suffisamment haut niveau pour qu'elle ne légitime pas, la remise en cause du statut des cheminots. J'espère enfin

est-ce une bonne idée, au moment où le gouvernement de Mme Theresa May, pourtant peu enclin à trouver quelque intérêt à la gestion publique, semble de plus en plus favorable à la renationalisation de certaines parties du réseau britannique dont les exploitants sont en grande difficulté financière Est-ce vraiment une bonne idée, sachant que c'est précisément la logique d'ouverture à la concurrence qui, voilà vingt ans, a conduit à la création de Réseau ferré de France, première mouture de SNCF Réseau, produit juridique de la séparation entre infrastructures et exploitation, devenu réceptacle d'une dette ferroviaire progressant de manière inexorable ? Il faudra bien, un jour, que les technocrates européens comprennent que la logique de marché n'a pas véritablement sa place dans un secteur ferroviaire où l'intensité capitalistique et la faiblesse des rendements attendus limitent, par principe, le nombre des tickets d'entrée dans le grand bal de la concurrence libre et non faussée ! D'ailleurs, la SNCF doit être le premier opérateur non britannique sur le marché ferroviaire outre-Manche, suivie à brève distance par Transdev, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, et l'on se souviendra que c'est la Deutsche Bahn qui est venue concurrencer, par filiale interposée, la SNCF en France pour le transport du fret. Cette situation d'oligopole obligé, si l'on peut dire, n'exclut évidemment pas de recourir à l'argent public quand il s'agit d'équilibrer les comptes. Ni le contribuable ni l'usager des transports n'ont donc grand-chose à attendre de cette ouverture à la concurrence. Quant à ceux qui en attendent des effets bénéfiques pour l'aménagement du territoire, ils seront sans doute quelque peu déçus, puisque le syndrome de réduction des dessertes frappant les de l'ex-République démocratique allemande, par exemple, risque fort de trouver sa traduction hexagonale.

d'une ouverture à la concurrence pour l'ensemble du réseau ferroviaire national. Il est vrai que le réseau francilien est spécifique,

nous avons un désaccord de fond : une délégation de service public à un opérateur privé, ce n'est pas la même chose qu'une délégation de service public à un opérateur public national, voire à deux opérateurs nationaux aux missions complémentaires, comme la RATP et la SNCF. Je vais prendre un exemple précis. Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice de transport en Île-de-France, souhaite confier à une filiale privée de la RATP la mise en exploitation de la future ligne du tramway T9,

et je n'y reviendrai pas -, y compris pour les passagers, notamment une baisse de la qualité de service. Cette ouverture à la concurrence se traduira par l'intervention d'une multitude de sociétés privées, dont le principal souci sera non pas le service rendu à égalité à chacune et à chacun, mais la recherche de la rentabilité maximale. Ce n'est pas

l'on se bat pour qu'il n'y ait plus de « petits gris » en Seine-et-Marne ! Cela fait vingt ans que l'on dit que le service est sursaturé ! Cela fait vingt ans que l'on essaie de faire en sorte que la ligne 13 fonctionne ! Cela fait vingt ans que l'on souligne que le système des RER a été fait de manière folle, avec des interconnexions qui n'en sont pas

Le scrutin est ouvert.

Outre l'opposition de notre groupe à l'ouverture du rail à la concurrence, dont on voit bien que même les Britanniques reviennent, l'idée même d'un échéancier pour les mises en concurrence nous interroge.

autre écueil tient au choix même de la ligne E. L'argument avancé en commission a été que le matériel y est plus récent- c'est vrai -, ce qui permet des taux de ponctualité et de régularité supérieurs.

situation. Il est proposé de permettre l'ouverture à la concurrence dès 2025 pour une ligne qui sera probablement en pleins travaux à cette date. De fait, si l'extension vers Nanterre-La Folie et Mantes-la-Jolie est censée être terminée en 2024,

des trains de la ligne P du Transilien vers Provins et Coulommiers et des TER Champagne-Ardenne. En toute logique, l'ouverture à la concurrence risque de surcharger des voies déjà saturées, au mépris de la qualité du service, mais aussi de la sécurité des passagers. Dernier problème, et non des moindres : l'extension vers l'Ouest parisien est une nécessité. En effet, la station Haussmann-Saint-Lazare n'a pas la capacité d'être un terminus, ce qui explique

si l'on ne veut rien reconnaître comme inconnu et nouveau, on a une pensée dogmatique, mais si l'on ne veut rien tenir pour connu et acquis, on ne peut avoir qu'une pensée inconsistante.

pourrait décider, à partir de 2025, d'ouvrir la ligne à la concurrence. Pour ma part, je fais confiance au STIF pour fixer le bon calendrier d'ouverture à la concurrence. Avis défavorable.

et mesure les nombreux désagréments qu'ils subissent. J'invite souvent mes collègues agriculteurs qui ne comprennent pas bien les attendus de ce débat à faire l'expérience physique d'un déplacement dans le RER B ou le